dernier, à zéro heure. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a été publiée. Cette candidature sera ratifiée

lors du scrutin n° 4 du 31 octobre 2017, portant sur l'ensemble de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la mission d'accueil des gens du voyage, Mmes Nathalie Delattre et Véronique Guillotin, MM. Stéphane Artano et Franck Menonville ont été déclarés comme ayant voté contre, alors qu'ils souhaitaient voter pour. Par ailleurs, Mme Josiane Costes et moi-même souhaitions nous abstenir. Ce sont, monsieur le président, de petits réglages de début de session Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur du Sénat, une délégation de cinq parlementaires de l'Assemblée fédérale suisse, conduite par M. Fathi Derder, conseiller national. Cette délégation est accompagnée par notre collègue Cyril Pellevat. La délégation est en France pour une visite d'étude, centrée autour de trois thèmes : les liaisons, en particulier ferroviaires, entre la France et la Suisse, ... Ah ... C'est un sujet, en effet. ... l'innovation, dans la perspective d'un renforcement de la coopération dans les domaines de la science, de la recherche et des transferts technologiques enfin, les conséquences du nouveau découpage des régions sur les relations avec la Suisse. La délégation s'est ainsi rendue hier après-midi au siège de la SNCF, à la Plaine Saint-Denis. Au Sénat, elle s'est entretenue avec les membres du groupe interparlementaire d'amitié France-Suisse et avec notre collègue Daniel Dubois, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, sur les crédits de la recherche. Le Sénat français entretient d'excellentes relations de confiance et d'amitié avec l'Assemblée fédérale suisse, qu'illustre l'organisation l'an passé, au Palais du Luxembourg, d'un grand colloque sur le cinq-centième anniversaire du Traité de Fribourg instaurant la « paix perpétuelle » entre la France et la Suisse. Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues du Parlement suisse la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, madame le rapporteur de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur de la commission du développement durable, saisie pour avis, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, chers amis, le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi que, à terme, à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, selon l'expression consacrée, et portant diverses dispositions relatives à l'énergie est l'une des pierres angulaires de la stratégie de la France pour lutter contre le changement climatique.

c'est un axe qui doit guider, orienter nos politiques publiques dans les décennies à venir.

la fenêtre d'opportunité dont l'Humanité, dans sa grande diversité, peut bénéficier pour empêcher cette irréversibilité est, c'est vrai, de plus en plus étroite

La France a été incontestablement dans le partage du diagnostic et dans la prise de conscience ; il faut lui reconnaître que, dans l'Accord de Paris, qui tient presque du miracle diplomatique, elle a permis l'établissement de cette feuille de route mais une feuille de route ne vaut pas succès et nous entrons maintenant dans la mise en oeuvre. Là aussi, nous devons être exemplaires. Le principe même de l'Accord de Paris est de créer une dynamique irréversible,

En rédigeant cette intervention, je pensais à cette phrase de Jean Monnet selon laquelle « les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise ». Nous sommes déjà dans la crise climatique, qui a frappé durement, ai-je besoin de le rappeler ?, les Caraïbes, où s'est rendu le Premier ministre- il nous en a fait un compte rendu il y a quelques instants en conseil des ministres et qui ne cessera hélas de nous rappeler à l'ordre. La démonstration qui en a été faite à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, qui nous a probablement plus touchés en raison de notre proximité géographique, citoyenne et culturelle, n'est qu'un sinistre échantillon de ce qui risque de se répéter dans un avenir proche. La tentation, face à la complexité de l'effort, que je ne sous-estime pas,

l'après-énergies fossiles, en devenant l'un des premiers pays à bannir de l'ensemble de son territoire la recherche de nouveaux gisements d'hydrocarbures, et à en limiter l'exploitation jusqu'à l'horizon 2040

les responsables, il faut faire preuve de cohérence. Je m'aperçois, je le dis sans procès d'intention, que, si tout le monde partage l'inquiétude et la volonté d'agir contre le changement climatique,

pour avoir une chance de gagner la bataille climatique, une chance de ne pas entrer dans ce phénomène irréversible, nous devons renoncer volontairement à exploiter 70 % à 80 % des réserves d'énergies fossiles que nous avons, facilement accessibles, sous nos pieds. Difficile de renoncer volontairement à une telle aubaine, tant nos sociétés ont été inféodées, associées aux énergies

et nous libérer progressivement mais irrévocablement de notre dépendance aux énergies fossiles. Avec l'adoption du plan Climat, la France a déjà fait sien l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Vous le savez, ce plan décline un certain nombre de moyens et d'actions permettant de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. au passage une petite réflexion supplémentaire. Si l'impératif climatique ne nous précipitait pas dès maintenant dans l'obligation de sortir des énergies fossiles,

C'est à cette condition que nos politiques publiques seront en cohérence avec la loi de transition énergétique, qui prévoit, je le rappelle, d'atteindre 32 % d'énergies renouvelables en 2030

J'ai écrit au commissaire européen chargé des transports pour l'encourager à adopter une réglementation plus ambitieuse pour l'Union en 2025 et en 2030.

D'abord, je ne pense pas qu'elle soit pénalisante, car elle nous permettra de nous mettre le plus rapidement possible en ordre de marche pour bénéficier des opportunités de cette transition énergétique. Ensuite, je ne peux pas me priver

; ce que Paris commence, l'Europe le continue. » J'espère qu'il en ira de même avec ces objectifs. Ce projet de loi s'inscrit donc dans une logique d'ensemble qui vise à nous redonner, c'est très important, notre liberté de choix en matière de politique énergétique. Cette logique d'ensemble s'appuie sur deux piliers. Le premier consiste à réduire la consommation d'énergies fossiles, c'est la clef de notre indépendance.

de la géopolitique mondiale. Notre dépendance aux hydrocarbures nous place aussi dans une situation de dépendance vis-à-vis des pays producteurs.

jamais très éloignées des sources de conflits auxquels nous avons assisté depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai tendance à penser que, en nous libérant de cette dépendance, nous nous soustrairons à autant de sources de conflits à venir. C'est pourquoi je considère ce projet de loi comme un pilier d'une stratégie beaucoup plus globale, qui vise à rendre la France indépendante et autonome sur le plan énergétique. Cet objectif fait sens. Il est ambitieux,

doit nous emmener vers une France peut-être pas exclusivement- l'avenir le dira -, mais majoritairement tournée vers les énergies renouvelables,

doit viser à faire de notre pays un pionnier des énergies propres, dans le domaine du stockage, mais aussi dans celui de l'hydrogène. Nos petites, moyennes et grandes entreprises nos industries couvrant l'ensemble de ces domaines, je suis intimement convaincu que nous pouvons également créer de nombreux emplois à l'occasion de cette transition. avec ce projet de loi, le Gouvernement vous propose tout simplement d'aligner enfin notre droit avec nos objectifs de lutte contre le changement climatique, dans un souci de cohérence. Jusque-là,

ministre, j'ai moi-même découvert cette situation où prévalait un droit inadapté aux enjeux de notre siècle, où le droit de suite régnait en maître et empêchait le Gouvernement de refuser tout nouveau permis, alors même que nous savions que c'était contraire à nos objectifs de lutte contre le changement climatique. Je veux maintenant vous préciser rapidement ce qu'est la philosophie du Gouvernement, pour que cette transition puisse être assumée. Se pose d'abord la question des entreprises, des filières industrielles et des emplois.

avons d'ores et déjà commencé à dialoguer avec les acteurs qui s'y préparent, pour identifier les compétences qui vont devoir se transformer et, dans le même temps, appréhender les reconversions possibles. ne doute absolument pas que les énergies renouvelables puissent offrir des solutions de reconversion intéressantes, par exemple avec la géothermie.

avec les territoires qui seront concernés, pour que leur avenir ne dépende plus de la seule exploitation des énergies fossiles, mais s'appuie bien sur une diversité de ressources et d'activités. En fait, tout bien considéré, ce projet de loi ne fait qu'accélérer un rythme normal, qui est celui de l'exploitation des ressources naturelles : il y a toujours eu des gisements qui s'épuisaient et des exploitations qui s'arrêtaient.

doivent présenter une certaine souplesse pour pouvoir s'adapter à chacun des cas, mais ils reposeront évidemment sur une mobilisation interministérielle des services nationaux, nationaux, mais aussi, et surtout, territoriaux de l'État, avec l'aide de l'ensemble de nos opérateurs. Ce sont environ 3 500 emplois qu'il faudra réinventer d'ici à 2040.

et crée lui aussi, chaque année, de nombreux emplois, lesquels sont répartis de manière assez équitable sur l'ensemble du territoire. J'en profite d'ailleurs pour préciser que le Gouvernement a déposé, à l'Assemblée nationale, amendement, qui a été adopté, visant à simplifier le raccordement des installations d'énergies renouvelables en mer. Mais ce projet de loi est aussi une partie de notre réponse à ceux qui, notamment de l'autre côté de l'Atlantique,

si les mots ont un sens, si les rapports scientifiques en ont un, c'est bien cela qui est en jeu. C'est bien pour cela que, au-delà des différences culturelles, politiques, économiques, il serait presque indigne

mis à mal par l'effet domino des conséquences des changements climatiques. Ce projet de loi comporte aussi plusieurs dispositions

problème d'approvisionnement. Ainsi, les articles 4 et 5 du projet de loi vont permettre d'engager, et c'est très important, une réforme du stockage souterrain de gaz naturel, pour à la fois améliorer notre système de stockage et mieux le réguler, préciser les compétences de la Commission de régulation de l'énergie et favoriser une concurrence juste et, surtout, sans surrémunération de certains acteurs.

La seconde directive prévoit la réduction des émissions de certains polluants de l'air, toujours avec ce même souci de protéger les Français et la planète.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, en interdisant une production nationale qui couvre à peine 1 % de nos besoins en pétrole et 0,1 % en gaz, le Gouvernement a choisi le symbole au détriment de l'efficacité. Or, si la politique est parfois faite de symboles, les symboles ne suffisent pas à faire une politique. En premier lieu, il n'est pas question de contester l'urgence à agir pour le climat. D'ailleurs, sur ce sujet, le Sénat, notre commission en particulier, a prouvé sa détermination. Je rappelle que c'est grâce au soutien de notre commission qu'a été fixée une trajectoire ambitieuse de hausse de la taxe carbone dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. C'est encore le souci du climat qui a guidé notre défense d'un mix de production électrique décarboné reposant sur ses deux pieds, le nucléaire et les énergies renouvelables. Et, chaque fois que notre commission a dû se prononcer sur des textes européens, elle a plaidé pour une tarification la plus incitative possible du carbone. Sur ces questions, le Sénat a toujours défendu une vision à la fois ambitieuse et pragmatique. Or, où est le pragmatisme dans ce texte, dont le Gouvernement insiste sur la portée éminemment symbolique, le caractère pionnier et l'effet d'entraînement recherché sur d'autres pays ? Et qui peut raisonnablement imaginer que les grands pays producteurs d'hydrocarbures renonceront à leur rente pétrolière pour suivre l'exemple français, bien qu'ils soient pour la plupart signataires de l'Accord de Paris ? Une autre voie était possible pour agir sur le climat. Elle consistait à traiter le problème à la racine, c'est-à-dire par la consommation. Les hydrocarbures représentent encore plus des trois quarts de notre consommation énergétique finale. Dès lors, comment atteindre l'objectif d'une baisse de la consommation des énergies fossiles de 30 % en 2030 ? C'est la question à laquelle devrait prioritairement répondre le Gouvernement. Les pistes sont du reste nombreuses, bien qu'elles soient plus difficiles à mettre en oeuvre et plus coûteuses, au moins à court terme, qu'une interdiction de la production nationale, qui fait office de paravent bien commode. Il faudrait, en particulier, « muscler » les dispositifs d'aide à la conversion des véhicules, développer de nouvelles solutions de mobilité, relancer le transport ferroviaire, maritime et fluvial de marchandises, renforcer les aides à la rénovation thermique des bâtiments plutôt que de tenter de les diminuer. Derrière le symbole de l'interdiction, il y a surtout une réalité économique, sociale, industrielle et environnementale que l'on ne saurait ignorer, celle des 1 500 emplois directs et 4 000 emplois indirects de l'exploration-production sur le territoire national qui vont disparaître sans que la question de la reconversion soit abordée autrement que par la promesse d'un rapport et par l'annonce de « contrats de transition écologique et solidaire » dont le contenu comme les moyens restent à préciser. Au-delà de ces conséquences immédiates, on pressent déjà une perte d'attractivité auprès des jeunes, qui n'iront pas vers ces métiers, et une dégradation de l'image de la France aux yeux des investisseurs étrangers. Certes, la logique d'une interdiction à l'échelle nationale aurait pu se justifier si elle contribuait véritablement à lutter contre le réchauffement climatique. Or, en remplaçant une production nationale, même limitée, par des hydrocarbures importés par voie terrestre ou maritime et parfois produits en usant de techniques moins respectueuses de l'environnement, on dégrade notre bilan carbone plutôt qu'on ne l'améliore, puisque l'empreinte carbone du pétrole importé serait au moins trois fois supérieure à celle du pétrole produit localement. Le Gouvernement objecte que, en raison de la baisse supposée de la consommation, une telle substitution n'aura pas lieu, puisque le 1 % de la consommation couvert par la production nationale aura disparu. il restera toujours une part de la consommation que l'on aurait pu satisfaire par la production nationale, sauf à supposer une consommation nulle, mais ce n'est pas demain la veille.

celui d'équilibrer le texte, en préservant la recherche pour ne pas insulter l'avenir, en limitant l'atteinte aux droits acquis pour que l'État tienne sa parole et, au passage, pour qu'il n'ait pas à payer d'indemnisations très importantes et, enfin, en autorisant les usages vertueux dont il serait dommage de se priver par dogmatisme. de préserver la recherche, nous avons introduit une dérogation pour la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du sous-sol, de surveillance ou de prévention des risques miniers. de limiter l'atteinte aux droits acquis, nous avons prévu les « mesures transitoires plus substantielles » suggérées par le Conseil d'État pour traiter les demandes en cours d'instruction, tout en préservant le principe d'une interdiction à l'horizon 2040. La loi ne s'appliquera qu'aux demandes déposées après le 6 juillet 2017, qui est la date de présentation du plan Climat, afin d'éviter tout effet d'aubaine, à l'exception de l'encadrement du droit de suite qui, lui, vaudra y compris pour le passé. Les concessions qui pourraient en résulter ne pourront donc excéder le 1 janvier 2040. J'ajoute que, même dans l'hypothèse où la quarantaine de demandes d'octroi de permis concernées serait accordée, dès lors que, statistiquement, un permis de recherche sur dix aboutit à une exploitation, il ne serait question que de quatre ou cinq concessions au plus, et encore celles-ci devraient-elles cesser en 2040. J'y insiste, il s'agirait non pas d'attribuer de « nouvelles concessions », mais uniquement de respecter les demandes déjà déposées, que l'administration se refuse à traiter depuis des années parce qu'elle serait contrainte d'y faire droit en application du code minier actuel. Enfin, notre commission a autorisé les usages vertueux des hydrocarbures en étendant une dérogation déjà ajoutée à l'Assemblée nationale et en créant une nouvelle dérogation. En effet, pour permettre la poursuite de l'exploitation du soufre dans le bassin de Lacq, nos collègues députés ont autorisé l'exploitation des hydrocarbures dits « connexes Mais cette dérogation, pensée uniquement pour le gaz de Lacq, ne trouvait pas à s'appliquer aux hydrocarbures liquides connexes, dont la situation est pourtant comparable et qui contribuent à une valorisation locale de nos ressources. Deux exemples illustrent l'intérêt d'une telle exception : l'exploitation de pétrole permet déjà de chauffer gratuitement, à Parentis-en-Born, une dizaine d'hectares de serres de tomates et, dans le bassin d'Arcachon, les 450 logements que comportera à terme un écoquartier, grâce aux calories récupérées de l'eau issue du processus de production du pétrole. Sans valorisation du pétrole, cette activité de production de chaleur devrait cesser, faute de modèle économique, et de tels projets ne pourraient pas être développés à l'avenir. Nous avons donc adapté la dérogation pour couvrir tous ces cas. La seconde dérogation concerne les hydrocarbures destinés à un usage non énergétique dont l'utilisation finale du produit n'émet pas de gaz à effet de serre, puisqu'il n'y a pas de combustion. Les exemples de débouchés sont très nombreux : bitumes, lubrifiants, cires, colles, textiles synthétiques ou matières plastiques, autant de produits dont nous aurons évidemment encore besoin en 2040. Ces hydrocarbures produits localement viendront alimenter nos filières nationales, qui, sans cela, devraient recourir à des importations. Pour finir sur le volet « hydrocarbures », j'indiquerai simplement que notre commission a fait en sorte que l'encadrement du droit de suite préserve la rentabilité de l'activité. Enfin, elle n'a pas souhaité rouvrir le débat sur l'interdiction des techniques dites « non conventionnelles J'aborderai brièvement deux autres mesures importantes du texte. La première est la réforme du stockage souterrain du gaz naturel, sujet sur lequel le Gouvernement avait déjà été habilité à légiférer, mais n'avait pu aboutir dans le délai imparti. Compte tenu de l'urgence de la réforme et de son état d'avancement, notre commission a préféré l'inscrire dans la loi plutôt que de renvoyer à une nouvelle ordonnance. Je vous proposerai simplement quelques derniers ajustements techniques. La seconde mesure importante a été introduite à l'Assemblée nationale par voie d'amendement gouvernemental, alors que son lien avec le texte initial est loin d'être avéré. Elle vise à réformer les conditions de raccordement des énergies renouvelables en mer. En s'inspirant du modèle en vigueur dans les pays nordiques, qui a prouvé son efficacité, elle devrait permettre de réduire les délais de réalisation ainsi que les coûts de soutien pour la collectivité. Aussi, malgré nos réserves sur la forme, nous approuvons la réforme sur le fond. Nous sommes simplement allés au bout de sa logique en étendant les cas d'indemnisation possibles du producteur dans l'hypothèse d'une indisponibilité du raccordement. Enfin, en matière de distribution d'électricité, notre commission a souhaité mieux encadrer la notion de réseaux intérieurs créée à l'Assemblée nationale, pour sécuriser le monopole de la distribution publique et préserver la péréquation tarifaire, à laquelle nous sommes tous ici très attachés. sont, mes chers collègues, les principaux apports de notre commission. J'ajouterai, pour terminer, que l'examen en séance sera l'occasion de traiter un sujet sur lequel nombre d'entre vous ont été sensibilisés : je veux parler de la concurrence déloyale de certains biocarburants importés et du danger qu'elle représente, à très court terme, pour la filière française. Après analyse, il nous semble que l'urgence de la situation justifie qu'un dispositif transitoire de protection soit mis en place, en attendant que la plainte déposée devant la Commission européenne aboutisse.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, la France est mobilisée depuis plusieurs années pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de l'Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015, elle s'est engagée à agir pour contenir l'augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels. Lutter contre le réchauffement climatique nécessite avant tout de réduire notre consommation d'énergies fossiles, qui participent à hauteur de 70 % aux émissions de gaz à effet de serre en France. D'où notre regret, monsieur le ministre d'État, que le projet de loi que vous présentez ne comporte aucune mesure relative à la baisse de la consommation d'hydrocarbures et qu'il se limite à organiser la fin de la production de pétrole et de gaz sur le territoire national à l'horizon 2040. Monsieur le ministre d'État, vous parlez de course contre la montre pour lutter contre le réchauffement climatique, mais cette course doit s'organiser en équipe, en partenariat, en concertation avec les autres pays européens pour être efficace et pour dépasser la portée symbolique des mesures envisagées. Certes, vous avez plusieurs fois rappelé que ce texte ne devait pas être appréhendé seul et qu'il serait accompagné ultérieurement de mesures relatives à la réduction de la consommation énergétique et au développement des énergies renouvelables. Cependant, si nous comprenons l'urgence qu'il y a à réduire l'utilisation des énergies fossiles, la décision d'arrêter la production nationale d'hydrocarbures d'ici à 2040 nous paraît incohérente, pour deux raisons. Premièrement, 45 % de l'énergie finale consommée en France provient aujourd'hui du pétrole, contre 22 % pour l'électricité et 19 % pour le gaz. Bien sûr, il est souhaitable que la part du pétrole baisse, mais, selon certaines estimations, elle s'établira encore à 50 millions de tonnes en 2040, contre 75 millions de tonnes aujourd'hui. Deuxièmement, la décision de mettre fin à la production nationale d'hydrocarbures pourrait donc paradoxalement conduire à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, puisque la France devra substituer à cette production des importations d'hydrocarbures, qui génèrent beaucoup plus d'émissions de C02. En effet, selon certaines estimations, une tonne de pétrole produite en France émet trois fois moins de C02 qu'une tonne de pétrole importée. Nous risquons surtout de remplacer du pétrole et du gaz conventionnels par l'importation d'hydrocarbures non conventionnels, dont les modalités d'extraction et de transport sont dommageables pour l'environnement et fortement émettrices de gaz à effet de serre. Il s'agit d'un débat important. C'est aussi un débat d'actualité si l'on pense aux négociations entre l'Union européenne et le Canada sur l'accord économique et commercial global, le CETA. Dans son rapport au Premier ministre sur l'impact du CETA sur l'environnement, le climat et la santé, la commission indépendante mise en place rappelle que l'extraction et la consommation de pétrole brut issu des sables bitumineux canadiens génèrent un volume de gaz à effet de serre 41 % plus élevé que pour le pétrole classique. Ce projet de loi aurait dû, à notre sens, être assorti d'une réflexion quant à la mise en place d'un traitement différencié- par exemple, une taxation différenciée -des hydrocarbures importés en fonction du bilan carbone qu'ils présentent sur l'ensemble de leur cycle de vie. Malgré cette réserve de taille quant à la portée et aux effets du texte, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, saisie pour avis, n'a pas souhaité s'opposer à celui-ci, mais a cherché à en améliorer le contenu. La principale mesure du projet de loi vise à mettre progressivement fin à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures en France d'ici à 2040. Au regard du volume de la production nationale d'hydrocarbures, qui couvre 1 % de notre consommation annuelle, les effets de cette mesure seront doubles. Sur le plan de l'emploi et de l'activité, d'une part, les effets seront vraisemblablement limités. En termes d'investissements et d'innovation, d'autre part, cette mesure pourrait avoir un impact négatif sur l'ensemble de la filière pétrolière et gazière, en décourageant à l'avenir les investissements de recherche et de développement dans ces secteurs. Or ces investissements sont facteurs d'innovations, lesquelles profitent bien souvent à l'ensemble de la filière énergétique française. Continuer à investir dans la recherche et la connaissance de notre sous-sol est essentiel. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec ma collègue rapporteur de la commission des affaires économiques, Mme Élisabeth Lamure, prévoir explicitement que les activités de recherche sur les hydrocarbures réalisées sous contrôle public à des fins d'amélioration de la connaissance scientifique continueront à être autorisées. Bien entendu, ces activités de recherche ne pourront pas déboucher sur une exploitation des gisements. S'agissant des autres dispositions contenues dans le texte en matière d'énergie et d'environnement, je me limiterai à saluer la réforme des modalités de financement du raccordement des installations d'énergies renouvelables en mer prévue à l'article 5 Pour terminer, le projet de loi pose le problème de la vision globale de notre politique énergétique. En effet, on ne peut pas à la fois mettre fin à l'exploitation des énergies fossiles, développer les énergies renouvelables et réduire considérablement notre parc nucléaire sans remettre en cause notre indépendance énergétique et sans que la facture payée par les consommateurs augmente significativement. Nous ne sommes pas résignés, monsieur le ministre d'État, mais cette transition énergétique doit s'accompagner avant tout d'une révolution idéologique et philosophique qui doit dépasser largement les frontières françaises et européennes. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, telle est la position de notre commission sur ce projet de loi, dont vous avez compris qu'il ne nous satisfait qu'à moitié.

M. le ministre d'État, car il y a urgence et parce que le temps joue contre nous. Il n'est pas exagéré, en effet, de considérer que le sort du monde se joue en partie, de nos jours, dans la capacité des pays à se mobiliser contre le chamboulement climatique. Qui n'a pas encore constaté que les catastrophes climatiques que nous subissons partout sur la planète démontrent largement la vulnérabilité des sociétés humaines devant la force de la nature lorsqu'elles sont construites dans le déni de l'environnement Il n'y a que le président des États-Unis qui ne semble ni le constater ni le comprendre. Comme cela a déjà été cité, « pour la première fois, l'Humanité est en mesure d'anéantir sa propre espèce ». Voilà pourquoi il est devenu urgent de passer d'une société fondée sur une consommation abondante d'énergies fossiles à une société plus sobre et écologiquement plus responsable. C'est tout l'enjeu de la loi relative à la transition énergétique, c'est tout l'enjeu de ce projet de loi très volontariste, qui annonce clairement que la France s'engage dans la sortie des énergies fossiles, et c'est tout l'enjeu de l'Accord de Paris. Dans cet environnement mondial chamboulé au plan climatique, au plan climatique, dans ce monde plein d'incertitudes géopolitiques, il n'est pas de meilleure réponse aux enjeux écologiques, climatiques, économiques et sociaux. Et la France, par son exemplarité en ce domaine, peut contribuer à assurer le succès de l'ordre de mobilisation des nations contre le changement climatique. « Impossible ! », diront les

au-delà du symbolique, un texte de rupture qui bouscule les vieilles lunes et en termine avec le laisser-faire et le laisser-aller consistant à reporter les décisions difficiles sur les générations futures. Nous savons que le temps joue contre nous. Nous ne pouvons plus attendre, comme certains le pensent, qu'une main invisible- en l'occurrence, celle du marché -le fasse à notre place. Notre modèle énergétique n'est plus durable.

Il faut faire sauter le mur de l'argent et l'indifférence de certains propriétaires qui font obstacle au lancement des travaux. Reste, enfin, le chantier du développement des énergies renouvelables, où nous devons lever les freins de l'administration dans nos territoires.

Enfin, il faut aller dans le sens de la social-écologie, car, ne l'oublions pas, quand les conditions de vie se détériorent à cause d'un environnement dégradé, ce sont les plus faibles, les plus précaires qui en subissent les conséquences les plus graves. Le texte que vous nous proposez est à la fois audacieux et courageux.

de prévoir de solides mesures d'accompagnement et d'apporter des garanties concrètes aux territoires en transition. J'en termine en rappelant que, à l'issue des travaux en commission, nous nous sommes abstenus, non sans regret. Certains points d'achoppement sont apparus au travers des amendements adoptés : trop d'exceptions, trop de dérogations ont rompu l'équilibre du chapitre I. Nous défendrons donc plusieurs amendements visant à rétablir cet équilibre. Prenons garde de ne pas offrir un cheval de Troie à ceux qui veulent que rien ne change.

Nous approuvons notamment la transposition des directives sur les biocarburants et sur la réduction des polluants atmosphériques, à l'origine de milliers de morts. Nous espérons que le Sénat préservera toute sa force à votre projet de loi, monsieur le ministre d'État, que nous saluons. S'il est vrai que « le futur n'attend pas », alors il nous faut contribuer très vite à l'inventer. Gardons confiance, en cette période de COP23. Comme l'a dit Friedrich Hölderlin,

nous examinons aujourd'hui le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. C'est assurément un sujet d'importance pour notre pays au lendemain de l'accord climatique de Paris, sur lequel nous avons adopté une résolution à l'unanimité dans cet hémicycle, et à l'heure où Bonn accueille la COP23- nouvelle importante échéance internationale des négociations sur le changement climatique. Alors que les États-Unis ont décidé de se retirer de cet accord international sur la préservation de l'environnement, la France a plus que jamais un rôle de pilote. Pour préserver le consensus mondial, nous devons agir et faire preuve de courage en nous appliquant des règles exemplaires en matière de politique énergétique. Le projet de loi répond à cette ambition en réaffirmant nous objectifs de lutte contre le changement climatique tout en préservant nos mécanismes de sécurité d'approvisionnement. Vous l'avez souligné, monsieur le ministre d'État, ce texte est une pierre angulaire. Pour réussir le pari d'une limitation de l'augmentation des températures mondiales en deçà de 2° C, le pic d'émissions de gaz à effet de serre devra survenir, au plus tard, en 2020. Il faut donc aller vite et frapper fort en éliminant le plus rapidement possible l'usage des hydrocarbures. Le 30 octobre dernier, l'Organisation météorologique mondiale a publié son bulletin annuel, s'inquiétant d'une hausse dangereuse de la température et rappelant que, « la dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a trois à cinq millions d'années la température était de 2 à 3° C plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de dix à vingt mètres par rapport au niveau actuel » en raison de la fonte des nappes glaciaires. Mes chers collègues, le temps presse. En 2016, les températures de surface de la mer ont été les plus élevées jamais constatées. La hausse du niveau moyen de la mer s'est poursuivie, menaçant même certains pays océaniques de disparition totale. Ce phénomène, ne nous y trompons pas, touche également notre pays : sur la base d'une hausse du niveau des mers d'un mètre d'ici à 2100, la Camargue, l'estuaire de la Gironde seront profondément remodelés ; la vallée de l'Adour, la Vendée, une bonne partie du littoral de la Charente-Maritime et de la Somme, département qui m'est cher, seront submergées. Je ne parle pas de nos outre-mer, outre-mer, territoires ô combien solidaires des Îles Fidji qui président aujourd'hui la COP23. Faisons preuve de lucidité en prenant à bras-le-corps cette problématique et en nous engageant en faveur d'une neutralité carbone de notre pays. Le projet de loi va dans le bon sens : il met fin à l'exploitation d'énergies polluantes, conforte nos engagements en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques et de promotion des énergies vertes et il assure, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre d'État, à travers ses articles 4 et 5, la sécurité d'approvisionnement des Français pour protéger notre pays dans un monde où l'énergie sera, plus que jamais, un motif de conflit et de compétition internationale. Le groupe Les Indépendants- République et Territoires exprime par ma voix une réelle et sincère sensibilité sur ces problématiques climatiques. Il apporte donc son plein et entier soutien à cette initiative de révision de notre politique énergétique. », disait le président Chirac. Nous ne pouvons continuer de détourner le regard. Les travaux de l'Assemblée nationale ont saisi toute l'ampleur de ce texte pour l'avenir de notre planète et de notre pays.

; ce n'est pas rien, et il ne sera pas aisé de les supprimer -, l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste, au cas où une autre technique que la fracturation hydraulique pourrait être employée, ou l'information du consommateur sur le type de gaz fourni sont autant d'initiatives qui vont dans le bon sens.

le vote d'une dérogation pérenne pour la recherche réalisée sous contrôle public, à seule fin de connaissance géologique du sous-sol, de surveillance ou de prévention des risques miniers, pourrait aller dans le sens d'une forme de logique et de raison. Nous verrons, au cours du débat, comment les choses évoluent sur ce sujet.

choses seront difficiles. L'écologie n'est pas une contrainte, c'est une chance : l'inaction nous coûtera plus cher que l'action. Ces engagements ne font pas seulement de la France un pays pilote. Ils peuvent nous donner également une longueur d'avance dans la course commerciale et technologique demain. Ne cédons pas au fatalisme du « c'est trop difficile, on n'y arrivera jamais » ...

Monsieur le ministre d'État, vous nous aviez habitués à plus de talent pour trouver des solutions innovantes. Ce texte est purement dogmatique, c'est seulement un geste,

pour le maintien d'une filière que je continue de considérer comme environnementalement bonne, à savoir la filière nucléaire. Nous avons beaucoup de choses à faire bien plus utiles que de voter ce texte qui n'est qu'un geste. Mes chers collègues de la commission,

accorder à la commission ses aménagements et à faire en sorte que l'article 1 ne s'applique pas. Je vous remercie par avance, mes chers collègues, de nous soutenir.

Deux ans déjà se sont écoulés après l'accord historique de la COP21. N'oublions pas la barrière des 2 degrés qui va être difficile à tenir. Pour y parvenir, il est scientifiquement avéré que 80 % des ressources carbonées doivent rester dans le sous-sol.

Nous possédons déjà l'ensemble des technologies qui nous permettront de faire face aux enjeux : les énergies renouvelables et le développement des économies d'énergie,

à la transition énergétique, lequel portait aussi notre regard au-delà de la prochaine décennie, le groupe écologiste a introduit dans la stratégie bas-carbone la notion de 4 pour 1000 en agriculture, sur des bases scientifiques, devenue, lors de la COP21, un projet de recherche internationale. Quel est ce mécanisme ? Si nous parvenons à accroître le stockage naturel du carbone atmosphérique dans les sols de seulement 4 pour 1000, 0,4 % par an, nous pouvons stocker l'équivalent carbone des émissions totales annuelles de l'Humanité. Il s'agit d'un levier extrêmement puissant permettant d'atteindre plus rapidement l'inversion de la courbe des émissions pendant la phase de transition qui nous conduira vers une économie décarbonée. Je souhaitais rappeler cette avancée, qui permet de considérer l'agriculture comme un atout dans la lutte contre le changement climatique et non plus comme un problème. Cette initiative internationale, si elle est poursuivie et menée à son terme, doit permettre de concilier les objectifs

Certains ont pointé une incohérence : si nous devons nous priver d'exploiter nos propres ressources et que, dans le même temps, nous importons des combustibles fossiles dont le bilan carbone est moins bon, nous aurons

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, le projet de loi présenté devant notre assemblée vise à faire de la France une nation pionnière de la sortie des énergies fossiles. En pratique, ce texte permet aussi à l'État de sortir d'une forme de duplicité qui, s'agissant des demandes de permis, l'a souvent conduit à ne pas prendre de décisions, laissant les tribunaux le faire à sa place. Vous en conviendrez, la Guyane pâtit de cette duplicité depuis de nombreuses années. D'un côté, la majorité des demandes de permis restent sans réponse et, de l'autre, le décret censé transférer compétence en matière de titres miniers à la collectivité territoriale se fait attendre depuis sans que les condamnations prononcées par le Conseil d'État soient prises en compte. Dans ce contexte, vous comprendrez aisément que, en dépit d'une ambition partagée, mon collègue Georges Patient, sénateur de la Guyane, et moi-même portions des amendements visant à défendre les intérêts de notre territoire. En effet, comment expliquer aux Guyanais, en proie à des difficultés économiques et sociales profondes, qu'on leur interdit d'explorer leurs hydrocarbures, alors que chez nos voisins du Guyana, ExxonMobil annonce l'une des plus importantes découvertes d'hydrocarbures des dix dernières années. Imaginez un instant : si un tel projet venait à voir le jour en Guyane, comme le souhaite le géant américain, on parlerait d'un chiffre d'affaires potentiel de 100 milliards de dollars avec des retombées fiscales d'environ 420 millions de dollars par an pour la Guyane, et proches du milliard pour l'État. Je pose donc une première question, soulevée implicitement par le Conseil d'État lui-même : quelles contreparties réelles la Guyane et les outre-mer en général retirent-ils de ce texte, symbole qu'ils vont pourtant payer au prix fort ? Hormis Hormis quelques dispositions concernant les îles Wallis-et-Futuna, je regrette qu'aucune mesure d'adaptation ne soit prévue pour les territoires ultramarins, malgré leur faible contribution au réchauffement climatique et des difficultés économiques réelles. Certes, le Gouvernement a prolongé un permis d'exploration détenu par Total, avant de s'engager à prendre, d'ici à la fin de l'année, le décret tant attendu. Si je salue ces engagements, je crains néanmoins que nous soyons encore loin du compte, tant cette compétence ne sera plus qu'une coquille vide,

plutôt que de refuser expressément des demandes et d'avoir à les motiver ? À cet égard, le texte de la commission présente une avancée intéressante. En descendant massivement dans la rue, les Guyanais ont voulu faire savoir à toute la France qu'il ne peut y avoir, dans notre République, d'un côté opulence et puissance et, de l'autre, un sentiment d'abandon et de soumission. Au-delà de l'exaspération, je vous demande d'entendre l'aspiration profonde portée lors de cette mobilisation historique, celle de faire des Guyanais les premiers acteurs de leur développement. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, le mercredi 2 août dernier, l'Humanité avait consommé l'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en une année. Le coût de cette surconsommation récurrente est déjà visible : pénuries en eau, désertification, déforestation ou encore disparition d'espèces. Vivre à crédit ne peut être que provisoire, parce que la nature n'est pas un gisement dans lequel nous pouvons puiser indéfiniment. L'Accord de Paris a permis de définir une limite, celle des 2 degrés de hausse de température, comme un cap déterminant à ne pas dépasser pour éviter le déchaînement des éléments qui rendrait les conditions de vie difficiles et les changements irréversibles. Ouragans, inondations, sécheresses, incendies une séquence de catastrophes naturelles historiques, aggravées par le réchauffement climatique, frappe d'ores et déjà tous les continents. Pourtant, cette urgence climatique n'est pas partagée par tout le monde. Les climato-sceptiques remettent en cause les fondements du réchauffement climatique, quand certains grands groupes industriels ne se préoccupent souvent que de leur rentabilité financière à court terme, au détriment de la planète et de l'humain. Ce projet de loi interroge plus largement sur notre société de demain. En 2050, si nous n'agissons pas, l'ONU prévoit le déplacement de 150 millions de réfugiés climatiques. Comment ferons-nous, alors, pour accueillir des millions de femmes et d'hommes et faire société commune,

ce qu'il touche l'un des multiples aspects sur lesquels il faut agir pour sauver l'humain et la planète. Oui, l'action politique relève aussi du domaine symbolique ! Avec ce texte, nous pouvons envoyer un signal fort, celui d'une France qui prend ses responsabilités et qui, si elle saisit cette occasion, peut prendre la tête du combat inévitable contre le dérèglement climatique et pour la sauvegarde de notre planète. Dans ce cadre, il nous faut agir vite et fort, tant que la puissance publique et le pouvoir politique le peuvent encore. Si l'on peut regretter que ce projet de loi ne traite que de la production d'hydrocarbures sur notre territoire, laquelle ne représente que 1 % de notre consommation nationale, et qu'il ne définisse rien sur nos importations et nos exportations, nous pensons malgré tout qu'il

L'action isolée ne peut suffire, elle est comprise dans un modèle de société global. Le premier de ces actes consiste à refuser- c'est vital -le CETA, cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui va accroître la concurrence entre les secteurs agricoles, affaiblir les normes sanitaires et environnementales et entraver durablement nos politiques publiques. Absolument ! Le CETA, s'il venait à être mis en oeuvre, mettrait à bas le projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Oui, il faut le dire avec force : le CETA n'est pas climato-compatible et aucun garde-fou, monsieur le ministre d'État, ne pourra entraver sa dangerosité ! Je vous fais donc une proposition, ainsi qu'à tous mes collègues ici présents : malgré nos différentes sensibilités, nous oeuvrons autour de ce projet de loi dans un même objectif de préservation de la planète et nous oeuvrons, de manière générale et chacun à notre manière et avec nos idées, et avec nos idées, pour les Françaises et les Français. Pourquoi ne pas mettre alors entre les mains du peuple tous les éléments de ce traité de libre-échange, initier de grands débats publics et donner la parole à nos concitoyens par référendum, en acceptant, cette fois-ci, leur décision ? Ma deuxième proposition, c'est de systématiquement placer l'intérêt général, donc environnemental et social, avant les intérêts privés, partisans et financiers. Ce sera toujours le sens de nos amendements, car c'est ce qui anime nos combats politiques. Je prends un seul exemple. La date butoir de 2040 pour le renouvellement des concessions, déjà très tardive à notre goût, fait l'objet de multiples dérogations, notamment si le concessionnaire justifie justifie que la rémunération normale des capitaux n'est pas avérée. Une telle disposition fait primer la rentabilité sur l'exigence environnementale. Oui, monsieur le ministre d'État, le capitalisme financiarisé et mondialisé tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas, lui non plus, compatible avec les intérêts de l'humain et de la planète ! Il recherchera toujours la rentabilité immédiate et le profit à tout prix, au détriment de tout le reste. J'en viens donc à mon dernier point. Ce projet de loi, vous l'avez dit, doit s'accompagner d'autres projets de loi, notamment sur la place faite aux énergies renouvelables, l'objectif étant d'atteindre la part de 30 % du mix énergétique. Pour ce faire, il faut un investissement public massif

d'imaginer un moyen d'utiliser efficacement l'énergie du soleil, qui nous envoie chaque jour 8 000 fois nos besoins énergétiques. On va me dire que tout cela coûte cher ! Je fais donc une proposition

pour investir dans les énergies renouvelables, l'emploi et la formation ? Oui, il faut mobiliser l'argent qui dort tranquillement au soleil et ne profite qu'à quelques-uns, pour l'avenir de notre planète et pour l'Humanité ! Il faut donc des actes et, pour cela, il faut de la volonté politique. Je finis, comme c'est la coutume ici, nous fêtons aujourd'hui le centenaire de la révolution russe, permettez-moi de citer Lénine : « Là où il y a une volonté, il y a un chemin Croyez-le, monsieur le ministre d'État, il y a beaucoup de volonté au sein du groupe communiste républicain citoyen et écologiste pour trouver le chemin d'une société émancipée qui respecte l'homme et la planète

affiche les ambitions de la France et des cosignataires en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Je partage Puisque la COP21, qui a entériné ce traité international, a eu lieu en France, puisque notre pays a toujours été à l'avant-garde des défis planétaires et universels, il est légitime qu'il soit l'un des premiers à se montrer exemplaire. Seulement, monsieur le ministre d'État, la France ne doit pas être la seule ! Comme pour ce qui concerne l'application des normes européennes, pour lesquelles le Président de la République ne souhaite pas de surtransposition, nous ne devons pas être en décalage avec nos concurrents mondiaux.

C'est une intention ambitieuse, et il faut en passer par là. Cependant, nous devons assurer en droit la compétitivité de notre économie et de nos entreprises.

Je pense sincèrement, devant toutes ces préoccupations déterminantes pour l'avenir de la France, qu'il convient d'inscrire la réciprocité de la fin de l'exploitation des hydrocarbures dans la loi. Nous devons mettre un garde-fou nous permettant de prolonger l'exploitation si les autres pays ne nous suivent pas.

les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. C'est clair, notre droit constitutionnel exige que notre obligation soit tenue si les partenaires respectent leurs engagements. Vous dites que l'année 2040 est proche. Estimez-vous que nous ne consommerons plus d'hydrocarbures en 2040 ? Ou plutôt que nous n'aurons pas à en importer ? Comme vous, je le souhaite.

Nous le voyons au travers de vos références historiques, il a fallu une longue période de transition pour que l'homme, grâce à la technique, puisse battre le fer. Le symbole est fort, mais la temporalité est importante pour tendre vers une efficacité technologique. Car nous devons franchir des étapes.

De plus, en se privant de sa production nationale, la France favorisera plus encore l'importation de pétrole étranger, dont nous ne connaissons pas les conditions environnementales et sociétales d'extraction, contrairement à ce Nous bénéficions en effet d'un arsenal de normes et de contraintes permettant de protéger la biodiversité et les sols. Quel mauvais bilan pour le climat, monsieur le ministre d'État ! En effet, si l'on regarde le projet de loi que vous présentez avec une vision basique,

et leurs habitants. Dans la Marne- permettez-moi en cet instant d'associer à mon propos mes collègues Yves Détraigne et René-Paul Savary -, où nous avons des idées, mais aussi un peu de pétrole, les ressources de la redevance communale et départementale des mines représentent chaque année

Il s'agit de véritables écosystèmes industriels, qui se situent bien souvent dans des zones déjà touchées par la crise économique ou éloignées des zones d'emplois dynamiques.

Mais il faut trouver un équilibre dans le cadre d'un projet de loi, en prenant en compte un principe de réciprocité avec nos partenaires internationaux ; un principe de compétitivité des entreprises ; un principe d'écologie en consommant des hydrocarbures français, dont le bilan carbone est un principe de réalité s'agissant de la temporalité de la fin des hydrocarbures et des alternatives possibles. Nous sommes naturellement prêts à soutenir des mesures visant à lutter contre le réchauffement climatique. Mais telle n'est pas la question qui nous est posée aujourd'hui avec ce projet de loi. Nous disons « oui » à l'objectif, mais « non » à la méthode et ses conséquences. Vous le verrez, monsieur le ministre d'État, les amendements que certains d'entre nous ont déposés ne sont pas radicaux. Ils visent plutôt à conserver l'objectif d'une sortie du recours aux énergies fossiles, mais en atténuant les conséquences économiques et sociales néfastes pour nos territoires.

nous devons nous prononcer aujourd'hui sur des questions stratégiques pour notre ambition énergétique. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la méthode employée, car, si la majorité gouvernementale a changé, la méthode est restée la même et accuse plusieurs faiblesses dont nous ne pouvons nous satisfaire.

le coût de l'énergie pour les consommateurs et, surtout, notre projet de société, l'économie nationale et l'emploi. Cette méthode, c'est également celle des postures prescriptives et des objectifs chiffrés dépourvus de dimension économique et de vision stratégique.

Au contraire, je suis convaincu de la nécessité de ne pas adopter de posture et de croiser notre ambition en matière de transition énergétique à notre volonté dans le domaine économique, à notre vision de l'aménagement du territoire, à la valorisation de leur diversité, à une prise en compte des réalités sociales ou encore à notre conception du rôle de la France au sein de l'Union européenne et dans un monde qui, à l'horizon de 2050, comptera 9,5 milliards d'habitants.

je voudrais souligner non seulement l'ambition de ce texte, mais aussi sa cohérence avec ce qui a été entrepris par nos gouvernements au cours des dernières années.

et pose un premier jalon dans notre effort collectif de réduction de l'usage des énergies fossiles. Il fait également sienne la nécessité d'innover et d'investir dès aujourd'hui dans de nouveaux modes durables de production d'énergie, afin de contribuer à la transition énergétique. Ces objectifs sont en réalité, ne nous le cachons pas, un choix de société. Ils nous obligent par-delà les travées sur lesquelles nous siégeons et traduisent une vision résolument progressiste. La cause que vous défendez aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, à savoir la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures conventionnels comme non conventionnels, me tient d'autant plus à coeur que je suis élu de la Dordogne, un territoire potentiellement riche en ressources gazières et déjà ciblé par trois demandes de permis de recherches à Brive-la-Gaillarde, Cahors et Beaumont-de-Lomagne. La zone en question s'étend sur près de soixante-dix communes de mon département et englobe une importante partie de la vallée de la Dordogne, zone classée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO en 2012. Elle concerne également la vallée de la Vézère, riche en sites préhistoriques, comme celui de la grotte de Lascaux, et classée site remarquable. Ma vigilance sur ce sujet rejoint celle des nombreux collectifs formés sur le terrain, associations et élus locaux, qui se montrent inquiets s'agissant de l'avenir de ces permis. Dès lors, je l'ai dit, il y a tout lieu de saluer la cohérence de votre projet par rapport à l'action entreprise par François Hollande au cours son quinquennat, s'agissant tant des engagements pris au cours de la COP21 que des mesures inscrites en 2015 dans la loi relative à la transition énergétique. En outre, ce texte complète opportunément la loi de 2011 sur l'interdiction de la fracturation hydraulique, texte positif, mais source d'insécurité juridique. En effet, il n'interdisait nullement l'exploration et l'exploitation par recours à d'autres techniques que celle de la fracturation hydraulique, omission relevée très justement dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi

Nous espérons pouvoir vous convaincre, madame la rapporteur, que seule la définition que nous vous proposons, et qui n'est autre que celle de la proposition de loi de Nicole Bricq, permettra de poser un second verrou pour enterrer définitivement toute possibilité d'explorer ou d'exploiter des hydrocarbures non conventionnels. Car l'extraction du gaz de schiste sans fracturation hydraulique est déjà une réalité dans plusieurs pays, sans que les risques et dégâts environnementaux potentiels en soient pour autant diminués. Second point de vigilance que je souhaite mettre en avant aujourd'hui : les conséquences économiques et sociales de l'arrêt des activités déjà décrites d'ici à 2040. Ce texte, pour marcher sur ses deux jambes, un important volet de transition apportant le soutien nécessaire à la transformation et la mutation de l'activité des sites visés par l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures.

par mon collègue et ami Roland Courteau, c'est dans un état d'esprit constructif et résolument ambitieux que le groupe socialiste souhaite examiner ce projet de loi. Conscient de l'exigence qu'il porte, mais aussi de l'ampleur du défi posé,

le projet de loi que nous allons examiner est l'occasion pour moi d'aborder la question ô combien sensible de l'indépendance énergétique de la France. Vous l'avez rappelé devant nous, monsieur le ministre d'État,

-suppose de fermer non pas 17, mais 25 des 58 réacteurs du parc nucléaire français. Il suppose également de faire évoluer dans des délais très courts notre mix énergétique. Or, nous le savons, les énergies renouvelables ne pourront pas répondre à nos besoins à l'instar du nucléaire, sans rupture technologique s'agissant du stockage et du transport de l'électricité, ce qui ne semble pas de dessiner dans un horizon très court. Parallèlement, le texte vise à mettre fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire français, en fermant une soixantaine de gisements pétroliers et gaziers couvrant près de 1 % de la consommation nationale.

L'activité d'exploration et de production d'hydrocarbures a été au coeur de la constitution d'une filière pétrolière et gazière d'excellence, engendrant actuellement un chiffre d'affaires employant 64 000 personnes en France et faisant vivre quelques-uns de nos territoires. Ce texte aura pour conséquence de fragiliser une filière industrielle dans laquelle la France est en pointe, ainsi qu'un tissu économique composé d'entreprises de toutes tailles. Pour autant, ce texte n'aura pas pour conséquence de faire diminuer la consommation nationale d'hydrocarbures.

ce qui est tout à fait paradoxal, vous en conviendrez. Les travaux de la commission des affaires économiques ont permis de rendre ce texte plus réaliste. Je tiens à ce stade à saluer l'excellent travail des deux rapporteurs.

L'enjeu primordial de l'indépendance énergétique, c'est aussi la question de la survie des biocarburants français, aujourd'hui menacés à la suite d'une baisse importante des droits de douane européens. Le contexte dans lequel se trouve la filière française et européenne de biocarburants est, vous le savez, très alarmant. En septembre, l'Union européenne a pris la décision de réduire significativement les droits antidumping appliqués au biodiesel argentin. Telle est la concurrence déloyale qui va être installée grâce au gouvernement français, si rien n'est entrepris en l'état actuel. Une hausse massive des importations de ce carburant fait craindre des effets désastreux non seulement sur l'environnement, mais aussi sur un secteur de l'économie performant, qui verra sacrifiés les emplois qu'il génère, c'est-à-dire environ 20 000

Ce texte nous donne l'opportunité de prendre des mesures transitoires permettant de répondre à l'urgence de la situation, le temps que la Commission européenne se penche sur la question. J'aurai l'occasion d'y revenir pendant les débats, à l'occasion de la défense de deux amendements que j'ai déposés. Je proposerai ainsi de relever le niveau d'exigence en termes de durabilité, c'est-à-dire en termes d'émissions de gaz à effets de serre, soit pour les seuls biocarburants importés depuis un pays situé hors de l'Union européenne, soit pour tous les biocarburants importés,

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, nous avons tous dans un coin de la tête la date du 21 juillet 1969 et la célèbre formule de Neil Armstrong : « Un petit pas pour l'Homme, un grand bond pour l'Humanité. Comparaison n'est pas raison, certes, mais nous pouvons, sans ambages, affirmer que ce projet de loi que vous portez, monsieur le ministre d'État, est de la même veine. Vous l'avez dit devant les sénatrices et les sénateurs lors de votre audition, et l'avez répété aujourd'hui : il s'agit d'une loi pionnière, et nous espérons qu'elle fera contagion. L'esprit de cette loi est simple : prendre un chemin sans attendre que d'autres prennent l'initiative. Et chacun sait bien, vous l'avez dit, que, lorsque la France donne l'exemple, il arrive parfois que d'autres pays, d'Europe et d'ailleurs, suivent cet exemple. Ce projet de loi fait partie d'un tout, nous en sommes conscients, car nous savons pertinemment que les hydrocarbures extraits sur notre territoire représentent 1 % de notre consommation.

par la réduction de notre consommation, objectif incontournable partagé par les entreprises et les citoyens de ce pays, assortie du développement à grande échelle des énergies renouvelables. Il s'agit bien d'une loi pionnière, qui est en outre une loi de cohérence. C'est la cohérence qui nous permettra de gagner la bataille climatique Cette bataille a commencé depuis maintenant un certain temps ; nous savons qu'elle comptera plus de bénéficiaires que de perdants. La transition énergétique est une transition des modes de transport, des modes de production agricole, du logement : autant de champs d'emploi, d'innovation et de recherche très importants. La cohérence consiste aussi à accompagner cette loi de mesures de solidarité en direction des plus modestes. Le « paquet de solidarité climatique » prévu dans le projet de loi de finances que nous aurons l'occasion d'examiner prochainement comprend un certain nombre de dispositifs, notamment la prime à la reconversion pour des véhicules moins polluants, l'aide au remplacement des chaudières et, plus globalement, à la rénovation des bâtiments. Transition écologique et solidarité en direction des plus modestes sont bien l'alpha et l'oméga de la politique ambitieuse portée aujourd'hui par le Gouvernement ; nous ne pouvons évidemment que nous en réjouir. Cette loi n'a de sens que si elle entraîne les autres, et je suis certain que, dans les couloirs de la COP23, à Bonn, l'initiative française devrait être souvent évoquée ! N'ayons pas peur d'assumer cette transition écologique et faisons de cette dernière une chance pour nos territoires, en plaçant au coeur du réacteur, si vous me permettez cette image, la question des entreprises, des filières industrielles et des emplois. Le travail avec les territoires a déjà démarré. Il vise à identifier les compétences pour lancer la transition énergétique ambitieuse que nous appelons tous, ici, de nos voeux. Oui, les énergies renouvelables sont notre avenir, et nous avons l'impérieux devoir d'y consacrer des moyens, à la hauteur du mouvement engagé aujourd'hui à l'échelle du monde ! Avec ce projet de loi, nous donnons à notre pays une chance plus qu'une contrainte. Le texte comporte des dispositions qui permettent de répondre aux défis du climat, mais aussi à celui de la sécurité de l'approvisionnement énergétique que nous devons au consommateur ; d'autres mesures sont des transpositions de directives européennes. Ce dispositif est le premier étage d'une fusée qui doit nous conduire sereinement vers une transition énergétique partagée et ambitieuse. Nos collègues députés, en le votant, ont parfaitement intégré les grands enjeux qui sont devant nous. Le texte, Le texte, enrichi au cours des débats à l'Assemblée nationale, est parfaitement équilibré ; il concrétise bien les engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement. Nous souhaitons que notre assemblée Nous allons désormais entamer l'examen des amendements déposés ; nous serons évidemment particulièrement attentifs à ce que l'esprit initial du projet de loi ne soit pas remis en cause. Monsieur le ministre d'État, vous pouvez compter sur les sénateurs du groupe La République En Marche pour que nous fassions ensemble le bond de la transition énergétique, de la transition écologique.

nous oblige à ne pas baisser la garde et à faire le maximum. Et si je devais m'obstiner sur cet objectif, au risque de repousser la fermeture des centrales à charbon ou même de rouvrir des centrales thermiques pour parer aux risques d'approvisionnement,

qui disait : « Nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets dont nous continuons à adorer les causes. » D'une manière ou d'une autre, il faut que nous sortions des énergies fossiles !

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, chers collègues, ce projet de loi est essentiellement une modification fondamentale du code minier.

texte sur l'opportunité duquel je ne me prononcerai pas, mais qui sera applicable dans vingt-deux ans, après tout un tas de changements, je pense qu'il aurait été préférable de prendre en main la réforme d'un certain nombre d'aspects du code minier qui nécessitent de manière urgente

La séance est reprise. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

supprimé en commission des affaires économiques. L'article supprimé visait à ratifier l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier. Alors que le présent projet de loi procède à des modifications de la partie législative du code minier, nous considérons qu'il est utile de ratifier une ordonnance portant précisément sur la codification de celle-ci. Nous tenons à souligner que cet article 1 A

un projet de loi visant à réformer le code minier, et nous nous en félicitons. Nous sommes conscients qu'il sera nécessaire à cette occasion de corriger un ensemble d'erreurs à diverses adaptations. Comme vous l'avez vous-même souligné, en ratifiant cette ordonnance, il s'agit de permettre de mettre un terme à l'ambiguïté entourant le statut des articles du code minier issus de la recodification portée par l'ordonnance de 2011 et dont la légalité

« la ratifier brutalement risquerait de remettre en cause les dispositions adoptées ultérieurement » et que ce travail avait « vocation à être fait dans le cadre de la réforme du code minier ». Je souscris totalement à ces propos. C'est pourquoi j'ai proposé à la commission de supprimer l'article J'ajoute qu'il serait inconséquent d'autoriser la ratification d'une ordonnance sans la modifier tout en sachant que certaines dispositions devraient l'être. En outre, je ne crois pas que l'on grandisse le rôle du législateur en ratifiant à l'emporte-pièce,

minier issus de la recodification portée par l'ordonnance de 2011 et dont la légalité est malheureusement parfois encore remise en cause. Le Gouvernement souhaite le maintien de l'article dans le projet de loi. Je suis donc favorable à cet amendement.

une réforme du code minier pour ratifier une telle ordonnance ? J'ai l'impression qu'il serait préférable de ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. La parole est à M. Jean Louis Masson,

on empêche les gens qui pourraient attaquer telle ou telle disposition devant le Conseil d'État de le faire. Mais cela revient à reconnaître nous-mêmes que telle ou telle disposition figurant dans l'ordonnance n'est pas nécessairement conforme aux principes du droit

Son article 1, qui interdit l'obtention de titre minier au-delà de 2040, se veut un message clair sur l'urgence d'une transition énergétique et la fin d'une dépendance exclusive aux produits pétroliers. C'est un beau message pour nos enfants, qui attendent de nous des mesures courageuses. Je regrette cependant les dernières évolutions, qui ont rendu ce projet de loi trop timide. D'un symbole fort et attendu, nous dérivons vers des dispositions souvent floues et aléatoires. Il n'y a pas d'avenir dans la prospection de produits carbonés. Nous devons l'acter et concentrer la recherche vers d'autres ressources et d'autres pratiques plus vertueuses. Je parlais de dérives : alors qu'aucune nouvelle autorisation ne devait pouvoir être attribuée, de multiples exceptions ont été ajoutées au nom de la préservation des droits acquis, c'est-à-dire le droit des concessionnaires de faire de l'argent pour faire de l'argent, indépendamment de toute considération environnementale, écologique ou sanitaire. Le permis ou la concession pourront ainsi être octroyés ou prolongés jusqu'en 2040, contrairement à ce qui était prévu dans le projet initial. Il n'y a plus d'extinction progressive, puisque l'ensemble des concessions arriveront à échéance la même année, soit dans vingt-trois ans : Pis, des concessions pourront être octroyées au-delà de cette limite si les concessionnaires démontrent que la rentabilité, et non le seul équilibre économique, n'est pas avérée à cet horizon. De quel équilibre parle-t-on ? Le seul équilibre qui puisse s'entendre est celui de notre planète. Cet équilibre-là ne se monnaye pas. Des concessions nouvelles pourront également être octroyées dans le cadre du droit de suite, qui permet qu'un permis de recherches donne droit ensuite à un permis d'exploitation. titres de recherche en cours pourront donner lieu à autant de concessions et les soixante-deux concessions en cours de validité pourront être prolongées. Autant d'exceptions qui dénaturent ce projet de loi. Nous le regrettons profondément, car nous en partageons l'ambition première. Soyons courageux ! Osons tourner la page ; il le faut maintenant. Nous devons respecter nos engagements et donner l'exemple. La parole est à M. Fabien Gay,

Ainsi, de nouvelles règles sont définies, notamment l'interdiction de nouvelles concessions minières ou de nouveaux droits exclusifs de recherches après 2040. Ces objectifs, nous pouvons les juger audacieux ou non. Mais, de toute manière, soyons clairs, ils sont extrêmement fragiles avec la signature par le conseil de l'Union européenne du CETA et sa mise en oeuvre provisoire au 21 septembre dernier, le Président de la République ayant fait le choix de ne pas mettre son veto. Pourtant, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, les conséquences du CETA seront désastreuses. Ainsi, le CETA pourrait permettre de nouveaux investissements dans les sables bitumineux canadiens, qui non seulement augmenteraient les émissions de gaz à effet de serre, mais pourraient stimuler l'importation de ce pétrole très énergivore et peu écologique en Europe. Nous importerions donc un hydrocarbure dont la nocivité est pourtant avérée et reconnue. Par ailleurs, et plus fondamentalement, le mécanisme dit de cour d'investissement introduit par le CETA pourrait permettre aux entreprises de contester des politiques climatiques d'intérêt public si elles contreviennent à leurs intérêts. Ainsi, le CETA précise que peuvent être contestées les décisions des États qui enfreignent le « traitement juste et équitable », constituent une « expropriation indirecte » d'une entreprise ou frustrent leurs « attentes légitimes Le projet de loi que nous examinons entre très directement dans ce cadre, au nom des droits acquis. La seule manière de se prémunir contre ce type de procédures est de se mettre hors de portée de la libre interprétation des juges et d'exclure clairement certains secteurs du champ d'application du système d'arbitrage. C'est le cas, dans le CETA, pour toutes les politiques liées aux subventions ou à la stabilité financière, mais pas des politiques visant à réduire les gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'avait recommandé le Parlement européen en 2015. Nous le regrettons, car il est évident que les entreprises n'hésiteront aucunement à saisir le tribunal d'arbitrage pour faire condamner la France. Monsieur le ministre d'État, il est temps de prendre toutes nos responsabilités et de faire entendre une voix forte de la France, pour refuser la mise en oeuvre du CETA, qui vide de sa substance ce projet de loi.

j'espère que la COP23, à laquelle vous allez participer la semaine prochaine, permettra de faire en sorte qu'un certain nombre d'États nous rejoignent et partagent notre détermination à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures. Il n'y a qu'à cette condition que le texte proposé aujourd'hui, pour lequel nous avons, je le répète, un positif, pourra être vraiment

On veut prouver aux Français que nous arriverons dans notre pays à limiter la production de gaz à effet de serre en supprimant la production française d'hydrocarbures, qui représente 1 % de notre consommation.

les hydrocarbures français produisent trois fois moins de gaz à effet de serre, sont trois fois moins chargés en carbone que ceux que nous importons. Si l'on suit les prévisions du Gouvernement,

n° 58 rectifié . La commission des affaires économiques a introduit une nouvelle catégorie d'hydrocarbures- les hydrocarbures destinés à un usage non énergétique -, permettant d'élargir le champ des dérogations à l'arrêt de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures

En permettant que les dispositions de l'article 1 ne s'appliquent qu'aux hydrocarbures destinés à « un usage non énergétique », on stoppe l'ambition du projet de loi- l'arrêt l'arrêt définitif de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures -, en élargissant le champ des dérogations, qui pourraient se multiplier. Dans le même temps, on permet la poursuite de la recherche et de l'exploitation dans notre sous-sol d'hydrocarbures liquides ou gazeux, pour des usages non énergétiques. Par ailleurs, force est de le constater, le projet de loi prend déjà en compte des possibilités de reconversion des sites pour valoriser d'autres activités, comme le gaz sulfuré du site de Lacq ou d'autres énergies renouvelables. Or, à entendre certains, l'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures condamnerait la géothermie. À ce que je sache, les activités de géothermie ne font l'objet d'aucune interdiction En 2013, la ministre de l'écologie, Delphine Batho, a signé deux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques, qui ont été suivis de nombreuses autres demandes de titres d'exploration. Fin mars 2015, un fonds de garantie dénommé le GEODEEP a été créé pour encourager le développement de la géothermie. La fin de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures ne devrait donc pas se traduire par la remise en cause des activités de géothermie, largement soutenues en France. Nous pensons que les exceptions doivent demeurer limitées et être strictement encadrées ; elles ne doivent pas devenir la règle.

utilisés pour un usage non énergétique. Or le code minier ne prévoit pas la notion d'usage lorsqu'il délivre une autorisation d'extraction d'une substance. De notre point de vue, cette disposition serait donc très difficile à mettre en oeuvre. Par voie de conséquence, elle pourrait même détourner tout l'esprit du texte. Par ailleurs, au-delà des évolutions prévisibles vers une économie circulaire et vers des bioplastiques, bioplastiques, il serait nécessaire de faire préalablement le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour ces usages non énergétiques, qui, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas totalement nulles, loin de là.

les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes à un gisement de substances non énergétiques faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines. La commission des affaires économiques du Sénat a élargi cette dérogation à l'exploitation des hydrocarbures connexes à d'autres usages du sous-sol. Nous considérons que l'extension de la dérogation réduirait considérablement l'ambition première du projet de loi. Cet amendement vise donc à circonscrire la dérogation aux seules substances non énergétiques, à l'exclusion des autres usages du sous-sol.

Nous souhaitons en effet rétablir la rédaction adoptée par les députés, qui prévoyait des dérogations permettant de poursuivre l'exploitation de gisements de substances connexes non énergétiques contenues dans les hydrocarbures liquides ou gazeux. La rédaction adoptée à l'Assemblée nationale prévoyait que les hydrocarbures ainsi extraits seraient strictement limités à un usage local, sans pouvoir être injectés dans des réseaux de transport ou de liquéfaction. issue des travaux de l'Assemblée nationale donnait la possibilité aux titulaires d'une concession d'hydrocarbures exploitant un gisement connexe aux hydrocarbures, ou valorisant un produit non hydrocarbure- le soufre du site du site de Lacq, par exemple -, de faire une demande de conversion de sa concession d'hydrocarbures en concession portant sur une substance non énergétique. Dans ce cas, le titulaire du titre minier devait faire la démonstration à l'autorité administrative de la connexité des deux ressources et de la viabilité économique de l'exploitation du gisement de l'autre ressource. Les dérogations à l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures étaient donc strictement encadrées. Or la commission des affaires économiques a nettement élargi le champ des dérogations en permettant d'intégrer ce type d'hydrocarbures dans un processus industriel et en limitant aux seuls hydrocarbures gazeux la stricte valorisation locale. Le présent amendement vise à revenir sur l'extension des dérogations possibles et à maintenir un encadrement strict de ces dernières.

des hydrocarbures connexes aux seuls hydrocarbures gazeux. Il convient de limiter l'exploitation des hydrocarbures connexes, qu'ils soient liquides ou gazeux, à une valorisation strictement locale, afin de préserver l'esprit du projet de loi,

combustion et donc n'émet pas de gaz à effet de serre. Les exemples de débouchés sont très nombreux, je n'y reviendrai pas. Je rappelle seulement qu'en 2016 la pétrochimie a consommé, en France métropolitaine, environ 11 % de l'ensemble des produits pétroliers en tant que matière première. Le Gouvernement avance deux objections. La première est que le code minier n'examine pas l'usage d'une substance lorsqu'il en autorise l'extraction ; cette disposition serait par conséquent très difficile à mettre en oeuvre. oeuvre. Sur le premier argument, c'est une évidence : le code minier n'examine pas les usages tant que le législateur n'en décide pas autrement, ce que nous faisons ici. Quant à la difficulté pratique, elle est parfaitement surmontable. D'une part, il est des cas où l'usage non énergétique peut être attesté sans aucune difficulté en raison de la nature même de l'hydrocarbure ; c'est notamment le cas de certains champs pétroliers pour lesquels le brut est assez lourd et sera essentiellement dédié à la fabrication de bitumes. D'autre part, pour les cas où la nature de l'hydrocarbure n'en restreindrait pas l'usage à des finalités non énergétiques, une traçabilité pourrait être organisée sans difficulté par la filière, par exemple un système de certification ou de labellisation. La seconde objection du Gouvernement consiste, d'une part, à laisser penser que les progrès de l'économie circulaire et des bioplastiques permettraient de nous passer de tous les sous-produits du pétrole tous les sous-produits du pétrole à l'horizon de 2040, ce qui me paraît utopique, et, d'autre part, à plaider pour une évaluation préalable du bilan carbone de ces usages non énergétiques. Or ces usages ne sont pas plus émetteurs de gaz à effet de serre que d'autres activités de transformation industrielle. Dès lors, faudrait-il renoncer à toute activité industrielle ? La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements de l'amendement n° 42 rectifié confond plusieurs notions introduites ou clarifiées dans le texte de la commission. Son premier alinéa supprime l'une des références, mais une seule, aux hydrocarbures à finalité non énergétique, quand son deuxième rétablit en partie la rédaction

d'ouvrir la dérogation à des activités de géothermie. Je m'étonne, sur ce dernier point, que les auteurs de l'amendement ne soient pas favorables au développement de la géothermie. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement,

n° 59 rectifié . La commission des affaires économiques a prévu une dérogation à l'arrêt des activités de recherche sur les hydrocarbures. Nous nous interrogeons sur la réelle portée de ces dispositions. Force est de souligner que les dérogations précédentes introduites par la commission permettent déjà la poursuite des activités de recherche concernant « les hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique ». Permettre de poursuivre la recherche en présentant cela comme une rare exception fortement encadrée, au sens où cette recherche doit se réaliser sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers », nous laisse particulièrement perplexes. On nous présente les choses comme si l'arrêt de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures allait sonner la fin de la recherche scientifique en France. Mais cette recherche scientifique publique n'existe-t-elle pas déjà aujourd'hui ? Serait-elle le monopole des compagnies pétrolières ? Devrait-elle disparaître du fait de l'arrêt progressif, à l'horizon de 2040, de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures par ces mêmes compagnies ? Vous l'aurez compris, nous ne sommes absolument pas hostiles à la recherche, et à la recherche scientifique en particulier, évidemment. Mais nous nous interrogeons sur le sens et la portée de cette dérogation nouvelle. Qui plus est, comme cela est souligné dans l'objet de l'amendement du Gouvernement, identique au nôtre, « la recherche dans le domaine du sous-sol à des fins de connaissance géologique, de surveillance ou de prévention des risques miniers ne nécessite pas la délivrance de permis de recherches d'hydrocarbures. La délivrance d'autorisations de travaux à des fins de développement de la connaissance restera autorisée, indépendamment des dispositions de ce projet de loi ». Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer les dispositions introduites par la commission des affaires économiques, qui ne nous paraissent pas utiles.

Leurs missions couvrent largement la connaissance géologique et la compréhension des phénomènes liés au sol et au sous-sol. Ces entités interviennent en appui des politiques publiques.

de surveillance ou de prévention des risques miniers ne nécessite pas la délivrance de permis de recherches d'hydrocarbures. La délivrance d'autorisations de travaux à des fins de développement de la connaissance restera autorisée, indépendamment des dispositions de ce projet de loi., interdire la délivrance de nouveaux permis de recherches d'hydrocarbures, quelle que soit la technique utilisée

de « recherche sous contrôle public », dont le but est l'amélioration de la connaissance géologique des sous-sols et la prévention des risques miniers. Une telle rédaction ménage des intérêts divergents et laisse la porte ouverte à des activités de recherche privées dont la finalité pourrait être déguisée. Pour des raisons de clarté, nous lui préférons les termes de « recherche publique », afin de garantir que toute future activité de sondage des sous-sols du territoire national soit seulement guidée par les besoins de la science et l'intérêt général. Confier l'exclusivité de la recherche géologique à la puissance publique correspond parfaitement à la philosophie du présent projet de loi et permet d'éviter tout détournement de son objet. Nous pourrions faire le choix de supprimer cette disposition ; nous préférons l'encadrer.

qui pourraient contribuer au développement de filières d'avenir et accompagner la transition vers un nouveau modèle énergétique. La recherche ainsi autorisée ne pourra donner lieu ni à l'attribution d'une concession ni à l'utilisation des techniques dites « non conventionnelles

dans son objet comme dans ses modalités. Néanmoins, même si telle n'est pas votre intention, madame la rapporteur, nous craignons qu'une telle dérogation ne serve de cheval de Troie

permet au titulaire d'un permis d'exploration, dont la prospection est fructueuse, d'obtenir quasi automatiquement une concession pour exploiter son site, sans mise en concurrence ni autre procédure. Par cette disposition, le titulaire n'est donc pas soumis au dépôt d'un nouveau dossier complet auprès de l'autorité administrative. Dans les faits, ce droit ôte à la population locale toute possibilité de faire valoir son point de vue et à la puissance publique toute maîtrise des conditions d'exploitation du sous-sol. Cet article du code minier a été rédigé au XIX siècle et, de manière incompréhensible, n'a pas été modifié depuis lors. Il avait été imaginé à l'époque pour attirer les investisseurs, qui n'avaient alors rien à voir avec les gigantesques multinationales que nous connaissons aujourd'hui. Se rangeant à l'avis du Conseil d'État, le Gouvernement n'a pas souhaité encadrer ce droit dans la version initiale du projet de loi, ce que je regrette. Plus volontaire, l'Assemblée nationale a obligé le Gouvernement à faire un compromis en inscrivant dans la loi la date butoir de 2040 pour toutes les concessions en cours cours issues d'un droit de suite, sauf si les industriels prouvent qu'ils n'ont pas rentabilisé leur investissement. La commission des affaires économiques du Sénat est revenue en arrière en précisant que cette disposition ne s'appliquerait qu'aux permis accordés après le vote de la présente loi. Ainsi, les trente-trois détenteurs actuels de permis de recherches pourront obtenir leur concession comme si de rien n'était. Cette situation va à l'encontre de l'esprit même du présent projet de loi et elle est incompatible avec le respect des engagements de l'Accord de Paris. Nous proposons donc d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette disposition, que ce soit pour les permis de recherches en cours ou pour les permis futurs. Cette restriction est indispensable. Ne nous inquiétons pas d'une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les industriels. Nous considérons en effet que la Charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle, pourra être opposée à tout recours. Comme vous l'avez précisé, monsieur le ministre d'État, « le droit de suite règne en maître ». Il est temps d'en finir.

présent amendement n'est finalement que l'application législative de l'article 55 de la Constitution, que j'ai précédemment évoqué devant vous. S'il est important que la France soit le premier pays à prendre des mesures relatives à l'application de l'Accord de Paris sur le climat, je tiens à le redire, elle ne doit pas être la seule Afin de ne pas pénaliser la compétitivité de l'économie française et surtout de respecter la hiérarchie des normes en appliquant scrupuleusement notre Constitution,

conditionnons l'arrêt des activités de recherche et de production des hydrocarbures en France à l'application de l'Accord de Paris par les autres États signataires, comme le prévoit l'amendement

Vous ne pouvez pas imaginer combien cette initiative que nous allons prendre, si tant est que le présent texte garde son sens et son ambition, va nous aider.

dira que nous ne prenons pas beaucoup de risque à montrer l'exemple et que la France est plus arrogante que déterminante dans le processus.

ça, c'est sûr ! -, notamment au moment où une grande partie du monde subit les conséquences d'un phénomène qu'elle n'a pas provoqué

et rafleront toutes les opportunités économiques de la transition énergétique. Je dis seulement qu'il y a un avantage économique à se fixer des horizons à long terme, avec évidemment des points d'étape.

Ainsi, le texte vise à parvenir à la fin de l'exploitation des hydrocarbures à l'horizon de 2040. Pour ce faire, il prévoit l'arrêt de toutes les concessions en cours à cette date. Dans la réalité, les concessions dont l'échéance est plus tardive que 2040 pourront continuer leurs activités, puisque la loi n'est pas rétroactive. De plus, il existe une exception introduite par le texte pour les concessions qui n'auraient pas atteint leur « rémunération normale » en 2040, disposition que nous proposerons de supprimer au travers d'un prochain amendement. Alors qu'existent déjà ces exceptions qui fragilisent cette date butoir, curieusement, le projet de loi laisse la possibilité de prolonger toutes les concessions en cours dont l'échéance arrive à terme avant 2040 jusqu'à cette date. Il va sans dire que cette disposition sera utilisée par tous les titulaires desdites concessions, ou presque, pour continuer leur activité économique jusqu'à la dernière minute. Dans une optique de transition énergétique efficiente, il nous paraît opportun que le texte prévoie plutôt, comme cela était envisagé initialement, que les concessions actuelles ne pourraient être prolongées au-delà de leur échéance, et ce dès la publication de la présente loi.

Cette disposition permettrait un arrêt progressif entre 2018 et 2050, plutôt qu'un arrêt brutal des extractions d'hydrocarbures dans notre pays, tout en respectant les engagements contractés par l'État. Pour les chefs d'entreprise et leurs salariés, cela offrirait une visibilité accrue quant à l'échéance au-delà de laquelle ils devront avoir entamé une nécessaire transition. Nous rappelons une nouvelle fois qu'il est indispensable d'extraire et de consommer moins de 20 % des énergies carbonées encore présentes dans les sous-sols de la Terre pour parvenir à l'objectif de l'Accord de Paris.

autoriser le dépassement de l'échéance de 2040 si le titulaire de la concession démontre que cette limitation ne lui permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation. Si ce n'est pas cela, alors je souhaite bon courage à ces entreprises ! Par ailleurs, je voudrais soulever une question très importante à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans ce texte : dans le cas où un accord initial de concession dépasserait la date de 2040- je parle bien d'un accord écrit, validé et signé

est à M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement a pour objet de permettre aux régions ultramarines de délivrer de nouveaux permis d'exploitation en mer et de prolonger sans date butoir les concessions existantes.

et de leur très faible contribution au réchauffement climatique, alors même que la part des énergies renouvelables du mix énergétique dans ces régions est importante. Par exemple, en Guyane, les énergies renouvelables- photovoltaïque, hydraulique et biomasse -représentent 61 % de la production d'électricité locale.

des régions ultramarines. Vous connaissez la situation locale : cette région est très particulière et le sous-sol marin a un potentiel très intéressant- le Conseil d'État le savait lorsqu'il a rendu son avis. Dans l'ex-Guyane hollandaise, le Suriname, et dans la zone du Brésil située juste à côté, il est procédé à des explorations qui semblent vraiment intéressantes. Dans la Guyane anglaise, le Guyana,

donc forcément un potentiel très intéressant. Alors, monsieur le ministre d'État, je connais votre réponse : « J'ai été formidable avec la Guyane, j'ai autorisé le groupe Total à avoir une petite zone d'exploitation. »

quand il s'est rendu en Guyane il y a dix jours, s'est engagé pour que le processus entamé aille à son terme, c'est-à-dire que les permis d'exploration débouchent sur des permis d'exploitation. Dans le rapport de la commission, j'ai lu avec plaisir, madame la rapporteur, que vous laissiez entendre que cette interdiction d'exploration

un mix énergétique qui fait la part belle aux énergies renouvelables. Monsieur le ministre d'État, je vous demande de nous laisser cette opportunité de développement endogène de la Guyane, au moins jusqu'en 2040, la date butoir que vous avez vous-même choisie.

de la commission ? J'entends les arguments des auteurs des amendements consistant à dire qu'il serait absurde, au vu de la situation économique et sociale de ces territoires, de se priver d'exploiter des ressources dont la présence est très probable, au moins au large de la Guyane, et dont les retombées économiques pourraient être importantes. S'agissant de la Guyane, je rappellerai que, pour ce qui concerne les permis exclusifs de recherches valides ou pour lesquels une demande est en cours d'instruction, ces amendements seraient en réalité largement satisfaits. Comme vous le savez, le Gouvernement a déjà prolongé, par un arrêté du 14 septembre dernier, le permis « Guyane Maritime » détenu par Total, qui avait pris fin le 1 juin 2016 ; il court désormais jusqu'au 1 juin 2019. À l'issue de cette phase, Total pourra demander, si les réserves identifiées le justifient, l'attribution d'une concession, qui ne pourra lui être refusée en vertu du droit de suite. J'ajoute que la nouvelle rédaction de l'article 2 adoptée par la commission permettra également que deux autres permis portant sur deux autres zones au large de la Guyane-

Ainsi, en combinant la prolongation déjà accordée par le Gouvernement et le texte adopté par votre commission, plusieurs concessions d'hydrocarbures pourraient être accordées au large de la Guyane si le potentiel de réserves était confirmé. Pour

le permis « Guyane Maritime ». Pour le reste, permettez-moi de vous dire que si j'accordais, pour les raisons que vous évoquez et qui sont parfaitement nobles et légitimes, une dérogation à nos territoires ultramarins, alors que d'autres États océaniens s'imposent eux-mêmes la contrainte de ne pas utiliser les énergies fossiles pour aller directement vers les énergies renouvelables, je perdrais un certain nombre d'arguments. Je dis simplement que l'arrêt des activités de recherche et d'exploitation vaut dans toutes les zones de juridiction française,

Je le dis parce que c'est ainsi ! Le seul enjeu pour le lobby pétrolier, ce sont les permis d'exploitation de la Guyane. Jouer le développement des territoires ultramarins, qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, pour justifier que le lobby puisse encore un instant un instant toucher des dividendes et des recettes, ce n'est pas correct ! La réalité du monde, c'est cette souffrance-là. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui- c'est notre responsabilité de parlementaire -, c'est sortir d'une machine infernale qui va tout broyer.

quitte à ce que les Antilles soient balayées. Mais qu'on le fasse au nom des territoires ultramarins, même s'il y a des enjeux très forts de développement de la Guyane- je serai le premier à soutenir un développement durable de ce territoire -, ce n'est pas politiquement correct

dans les cas où « la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol » l'exigent. Nous partageons la volonté ici exprimée de renforcer l'encadrement des activités d'exploration et d'exploitation autorisées après l'entrée en vigueur de la loi et de limiter au maximum leur impact sur l'environnement local.

Aujourd'hui, nous le savons tous, le code minier est largement lacunaire dans ces domaines. Nous allons même plus loin, en transformant la faculté en obligation. Ainsi, pour chaque titre minier octroyé, l'administration se verrait dans l'obligation de réaliser un cahier des charges. en souhaitant que ce cahier des charges puisse mentionner l'interdiction du recours à certaines techniques et limiter les formations géologiques auquel le titre s'applique. Vous l'aurez compris, il s'agit de prendre en compte les avancées de l'article 3, qui élargit la définition des pratiques interdites en mettant fin à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels.

lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale et supprimée par notre commission des affaires économiques. Loin de représenter une nouvelle complexité administrative, la possibilité pour l'autorité administrative d'établir un cahier des charges précisant les prescriptions particulières nécessaires pour tenir compte de la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques constitue une avancée. En effet, cette disposition permet de renforcer l'encadrement

un cahier des charges, si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques l'exige, lors de la délivrance ou de la prolongation d'un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ne nous paraît pas être une mesure disproportionnée dans un domaine où, par définition, les activités sont risquées et peuvent avoir des impacts environnementaux importants. Il s'agit donc de faire oeuvre de prévention en renforçant l'encadrement des activités d'exploration et d'exploitation autorisées après l'entrée en vigueur de ce projet de loi. Ce cahier des charges permettra également de tenir compte, le cas échéant, du résultat

et que ses contours comme ses conséquences éventuelles sur la délivrance des titres n'avaient pas été explicités. Au surplus, les intérêts visés sont déjà protégés par le code minier, en particulier par la police des mines, et l'autorité compétente a déjà toute liberté pour arrêter les modalités d'instruction des titres, sans qu'il faille mobiliser pour cela un nouveau concept source de complexification administrative, au mieux, et d'insécurité juridique, au pire. Par ailleurs, nous avons considéré que, si cette notion devait perdurer, elle ne pourrait trouver à s'appliquer aux seuls hydrocarbures et devrait être examinée dans le cadre de la réforme du code minier annoncée pour le courant de l'année 2018.

qui a été débattue lors de l'examen de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement, en janvier dernier. Le Gouvernement partage les préoccupations relatives à la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques.

préciser certaines préoccupations, interdire certaines techniques, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s'applique, ou encore tenir compte des résultats d'une éventuelle procédure de participation du public. En somme, dans certains cas, un cahier des charges peut être très utile. être très utile. Je n'y vois pas forcément une complexité administrative, voire une insécurité juridique, mais plutôt une meilleure protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques. En ce domaine, ce n'est jamais trop

Le projet de loi définit un cadre nouveau pour la délivrance de titres d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures. En revanche, les procédures d'instruction et de gestion des titres restent identiques ; les règles prévues par le code minier et le code de l'environnement restent applicables. Afin de favoriser l'intelligibilité de la loi et de lever toute ambiguïté, le Conseil d'État a souhaité que cela soit indiqué explicitement.

ce qu'il fait par définition sauf dispositions expresses contraires. En l'espèce, la section 3 créée à l'article 1 déroge au code minier uniquement dans les limites et sous les réserves qu'elle prévoit. Au surplus, un tel rappel pourrait même s'avérer contre-productif, car rien ne démontre que la liste ainsi fixée soit exhaustive. Un doute pourrait alors naître sur l'application d'autres dispositions non citées bien qu'applicables. Enfin, le présent amendement ne vise pas à revenir exactement à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. Cela, au-delà de l'inutilité de l'exercice, en montre bien la difficulté : la loi de 2011 n'est plus mentionnée, alors même que la référence au code de l'environnement est étendue à l'ensemble du chapitre relatif aux procédures de participation du public. Encore une fois, tout ce à quoi la loi ne déroge pas continue, par définition, à s'appliquer. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

de poursuivre leur activité au-delà de 2040. Passons sur la notion très floue de « rémunération normale des capitaux immobilisés », qui ne veut déjà pas dire grand-chose en langage économique et ne veut strictement rien dire en langage juridique.

pouvons être certains que tous les titulaires de concessions tenteront d'utiliser cette exception pour poursuivre leur activité. Quel organisme public contrôlera la véracité de leur comptabilité ?

La date de 2040 est suffisamment lointaine, dans une perspective d'endiguement du réchauffement climatique, pour qu'on ne lui tolère aucune autre exception que celles que la loi ne peut pas corriger faute de rétroactivité. Enfin, si une entreprise ne parvient pas à réaliser de bénéfices sur une concession entre aujourd'hui et 2040, c'est que le gisement d'hydrocarbures concerné ne méritait pas d'être exploité. L'intérêt général n'a pas à souffrir des erreurs d'appréciation économique des entreprises ! La parole

a modifié les dispositions relatives à la limitation du droit de suite, d'une part, en les intégrant à l'article 1 du projet de loi et, d'autre part, en introduisant la notion de « rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités

par rapport au retour sur investissement des capitaux Dans la version du projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale, les concessions attribuées en application du droit de suite pouvaient exceptionnellement s'étendre au-delà du 1 janvier 2040 si le titulaire du permis exclusif de recherches démontrait que cela était nécessaire pour couvrir les coûts de recherche et d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre économique par l'exploitation du gisement ». Notre commission des affaires économiques a substitué à cette notion celle de « rémunération normale des capitaux immobilisés ». Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui permet de mieux limiter le recours au droit de suite, conformément à l'esprit du projet de loi.

attribuées en application du droit de suite pourrait dépasser l'échéance du 1 janvier 2040 uniquement si le titulaire démontrait qu'un tel raccourcissement l'empêcherait de couvrir les frais engagés et d'atteindre ainsi l'équilibre économique par l'exploitation du gisement découvert. Notre commission des affaires économiques, comme chacun le sait, a remplacé la notion d'« équilibre économique » par celle de « rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités ». Quant à nous, nous considérons que la notion d'« équilibre économique » est plus facile à appréhender d'un point de vue juridique que celle de

La rémunération considérée comme normale des mines d'exploitation d'hydrocarbures n'est pas la même selon que le prix du pétrole est faible ou élevé ; elle n'est pas la même lorsque ces mines conventionnelles sont concurrencées par des hydrocarbures de schiste elle est encore bien différente selon que l'on se place du point de vue des actionnaires, dont la rémunération est constituée de dividendes, ou de celui des entrepreneurs, qui sont rémunérés pour le risque qu'ils prennent par par ce qu'on peut appeler le profit. Enfin, et c'est sans doute aussi le but recherché, cette notion de « rémunération normale des capitaux » permettra à la fois

de cet amendement aurait paradoxalement pour effet de supprimer l'encadrement de ce droit tel qu'il a été introduit à l'Assemblée nationale et amendé par notre commission. En supprimant cet alinéa, cet amendement permettrait aux nouvelles concessions

dans la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. Notre commission a choisi de maintenir cet encadrement pour éviter que la durée d'une concession nouvelle puisse excéder le 1 janvier 2040. par ailleurs que la rédaction retenue par notre commission ne fait que revenir à l'esprit de la rédaction initiale, qui retenait la notion de « rentabilité normale » de l'activité. Nous préférons quant à nous l'expression de « rémunération normale », qui est plus usitée en droit, mais cela revient exactement au même.

et est déjà utilisée, dans le code de l'énergie, pour fixer le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité, des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et de gaz, et des tarifs d'achat du biométhane, ou encore pour dimensionner les appels d'offres à l'effacement électrique. C'est pourquoi nous vous

permettant de restreindre la possibilité de dépasser l'échéance de 2040 pour la durée de la première concession tout en respectant les exigences prévues en matière de droit de suite. Il s'agit donc d'encadrer le droit de suite dans le respect des principes constitutionnels tout en revenant à l'esprit même du projet de loi. Quel est l'avis de la